La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 2 août 2017 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ?

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes saisis en nouvelle lecture

seule question de la réserve, même si celle-ci est devenue la mesure la plus emblématique et la plus discutée. D'autres dispositions, qui ont obtenu l'accord des deux assemblées, méritent toute notre attention comme celle de nos concitoyens.

et de la sanction infligée à ceux qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'impôt, du régime d'incompatibilité en matière d'activités de conseil et de représentants d'intérêts, lequel a d'ailleurs été renforcé hier en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, nationale, ou encore du droit de communication élargie pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sur tous ces points positifs, qui constituent de vrais progrès en termes éthiques,

N'est-ce pas en décalage par rapport à la volonté de recentrer les parlementaires autour de leurs fonctions constitutionnelles, qui consistent à voter la loi, à contrôler le Gouvernement et à évaluer les politiques publiques ? quel rapport les parlementaires doivent-ils entretenir avec le territoire où ils ont été élus ? J'ai entendu lors des différents débats, et encore hier à l'Assemblée nationale,

Ce n'est pas parce qu'un parlementaire ne peut plus donner de subventions qu'il est coupé de ceux qui l'ont élu, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils portent et de la réalité de ces territoires. Pour tout avouer, je trouve même qu'affirmer cela est une façon de nier le travail que les parlementaires accomplissent réellement sur le terrain. Une troisième question de principe se pose : doit-on conserver une pratique qui consiste, du moins je le pense, en un contournement des règles constitutionnelles par la voie coutumière ? La pratique de la réserve a certes l'apparence de la rigueur, puisque les parlementaires ne formulent que des propositions que le Gouvernement demeurerait libre de suivre Mais, en réalité, personne n'est dupe : les députés et les sénateurs sont bien les véritables ordonnateurs de ces dépenses. Je vais reprendre ici les mots d'un député, Jean-Louis Bourlanges, qui me semblent bien résumer notre débat. À l'occasion des échanges que nous avons eus à l'Assemblée nationale, il a affirmé que « la seule question qui nous divise est de savoir si nous, parlementaires, exerçons un pouvoir budgétaire collégial ou si nous bénéficions d'un démembrement de ce pouvoir, fût-il minime, qui nous permet d'exercer de façon individuelle un pouvoir fragmenté. Je réponds que nous sommes dépositaires de l'autorité budgétaire à titre collégial et que nous n'avons pas à nous ériger [ ...] en ordonnateurs fragmentés et particuliers. Chacun l'aura compris, la position du Gouvernement et celle qu'a réaffirmée hier l'Assemblée nationale reposent sur la clarté. Et cette exigence conduit à mettre fin à une pratique susceptible de créer de la confusion.

que la réserve permet de boucler des projets, de donner des moyens à des associations qui auraient peut-être du mal à s'en passer. Mais, sur ce point, les choses doivent être claires, dites et répétées : la suppression du mécanisme de la réserve parlementaire n'est aucunement un moyen inavoué de faire des économies sur le dos des collectivités territoriales ou des associations. Les questions financières liées à la préoccupation qui est la nôtre aujourd'hui devront être traitées au moment du débat budgétaire, et il appartiendra aux parlementaires d'exercer leurs prérogatives à l'automne, sur cette question comme sur les autres. Je note d'ailleurs que la commission des finances de l'Assemblée nationale a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait instituer un groupe de travail pour suivre la manière dont les crédits anciennement affectés à la réserve seront employés au profit des communes, des Français de l'étranger et des associations dans le cadre des instruments budgétaires de droit commun. J'ajoute que, si le Gouvernement avait eu l'intention cachée, en supprimant la réserve, de procéder à un tour de passe-passe budgétaire, il était plus simple pour lui d'opposer un refus aux propositions faites par les parlementaires lors de l'examen du prochain projet de loi de finances. Les deux rapporteurs l'ont reconnu en Le Gouvernement a donc préféré faire le choix de la clarté. Il a souhaité que la fin de la pratique de la réserve parlementaire soit débattue par le Parlement, ouvertement, publiquement, devant les Français. Et, de ce point de vue, je n'ose dire que nos espérances ont été totalement comblées

soit qu'il contraindrait le Gouvernement dans son droit d'amender les projets de loi de finances, soit, en sens inverse, qu'il ne serait pas normatif ou, enfin, que ce dispositif ne serait pas de nature organique. Sur ce sujet, j'invite chacun d'entre vous à relire l'avis du Conseil d'État, d'autant plus éclairant que le Gouvernement et l'Assemblée nationale s'en sont tenus à la rédaction proposée par celui-ci. Je cite cet avis, qui est

Un tel système dérogatoire au droit public financier n'étant pas formalisé, il devrait cesser d'exister par la seule volonté du Gouvernement de ne plus faire droit aux demandes des parlementaires, tant au stade de la discussion des projets de loi de finances que de l'exécution de ces lois. Toutefois, dès lors que la loi organique [ ...] du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a prévu la publication, en annexe au projet de loi de règlement, de la répartition des subventions attribuées au titre de la " réserve parlementaire ", la suppression de cette obligation de publicité figurant au sein de la loi -pourrait être complétée par une mention de l'interdiction de ce qui constitue juridiquement cette pratique, afin que le Parlement se prononce expressément sur la fin de cette pratique. sur la fin de cette pratique. Il s'agit en effet d'une des conditions dans lesquelles le Parlement vote les projets de loi de finances, conditions qui relèvent de la loi organique en vertu des articles 34 et 47 de la Constitution.

Il fallait aussi que la suppression de la réserve puisse être actée dans la loi organique. Le Gouvernement avait d'ailleurs envisagé de modifier la LOLF pour ce faire,

soit parce que le mécanisme violerait le droit d'amendement du Gouvernement soit, si tel n'était pas le cas, parce qu'il n'aurait alors aucune portée normative. À cette affirmation, je voudrais opposer- il s'agit là d'un débat juridique intéressant - les termes de l'article 34 de la Constitution, rappelés par le Conseil d'État, article qui dispose : « Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. » L'article 47 de la Constitution y fait écho, puisqu'il précise : « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. La loi organique doit donc fixer les conditions dans lesquelles sont examinés les projets de loi de finances. C'est le fondement constitutionnel de la LOLF ; c'est aussi celui de l'article 9 du présent projet de loi organique. Au surplus, et en tout état de cause, je rappelle que l'on pourrait également invoquer l'article 44 de la Constitution qui, depuis 2008, dispose que le droit d'amendement s'exerce par les parlementaires et le Gouvernement dans un « cadre déterminé par une loi organique.

Le Gouvernement, suivant strictement en cela le Conseil d'État, me semblait par conséquent bien fondé à insérer cette disposition de suppression de la réserve parlementaire dans une loi organique.

La normativité de ce dispositif ne fait donc aucun doute. Permettez-moi de considérer au passage que si cette disposition avait été dénuée de normativité, elle aurait sans doute suscité beaucoup moins de débats entre nous. La question posée est en réalité une question de principe. Certains estiment que la suppression de la réserve parlementaire met fin à une forme de clientélisme. Je n'utilise ni cet argument ni ce vocabulaire, car je ne souhaite pas aborder le sujet sous cet angle. Très bien ! Très bien ! Je crois simplement que cette pratique de la réserve crée de la confusion par rapport au rôle des parlementaires et que les Français souhaitent en cela, comme dans beaucoup d'autres domaines, de la clarté.

qui permettra d'engager un vaste mouvement de rénovation de nos pratiques politiques. Le vote de cette loi organique viendra couronner le travail accompli sur la loi ordinaire. Il sera la marque d'une volonté, celle de respecter les engagements pris devant les Français et, par cet acte de confiance, d'ouvrir la voie à un nouveau rapport à l'action politique.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame la vice-présidente de la commission des lois, mes chers collègues,

les membres du Gouvernement, sur la possibilité offerte au chef de l'État ou au Premier ministre de consulter la Haute Autorité pour la de personnalités pressenties pour entrer au Gouvernement, ou encore sur l'obligation pour le Gouvernement de publier dans les six mois un rapport sur le pantouflage.

une nouvelle étape dans la rupture du lien entre la représentation nationale et les territoires. J'apprécie la manière dont vous avez abordé la question,

députés et sénateurs se doivent d'être tout entier à leurs fonctions de législateur et d'autorité de contrôle de l'exécutif, et doivent en quelque sorte s'éloigner de toute responsabilité vis-à-vis des territoires qui sont à la racine de leur légitimité. Après l'interdiction du cumul de tout mandat avant la création d'un régime de représentation proportionnelle pour l'élection d'une partie au moins des députés, nous examinons aujourd'hui

d'intermédiaire entre la population et un État tout puissant serait un vestige du passé qu'il faudrait absolument éliminer.

qui vise à faire des représentants de la Nation de purs esprits, qui agiraient de manière aussi docile que possible vis-à-vis du parti politique dont ils sont les représentants, mais qui seraient en revanche libres de toute attache vis-à-vis du territoire qui les a désignés. Nous ne pouvons que combattre une telle approche, qui n'est d'ailleurs pas réaliste. D'une part, en tant que membres du Sénat, Sénat, nous représentons les collectivités territoriales de la République. D'autre part, nous entendons tout simplement, et je me permets de le dire avec une certaine gravité, défendre la démocratie.

l'expérience des réalités sans laquelle il n'y a pas de bonnes lois ni de capacité de contrôle indépendant du Gouvernement. Voilà pourquoi nous voulons combattre l'instauration d'un nouveau régime de démocratie d'opinion, ouverte à tous les vents et qui serait, un jour, balayée par les vents mauvais de l'extrémisme. Très bien ! La démocratie s'enracine dans la vie des territoires. Ce sont ces racines que l'on est en train de couper Je suis contrarié par l'hypocrisie qui est à l'oeuvre dans ce débat. On n'ose même plus reprocher

que l'accusation de clientélisme, dont il est aisé de faire justice, puisque la réserve est égale, transparente et accessible à toutes les communes, comme le Gouvernement, lui-même,

S'ajoutant à de nombreuses mesures récemment prises, et qui montrent la médiocre considération accordée aux collectivités territoriales par le Gouvernement, cette nouvelle disposition ne peut que susciter notre opposition tout à fait radicale.

pour faire en sorte que les collectivités territoriales ne soient pas les grandes oubliées de la nouvelle République que vous êtes en train de construire ! La parole est

utilement distribués à travers le mécanisme de la réserve continueraient à bénéficier aux mêmes fins d'intérêt public, qu'il s'agisse du soutien aux associations,

on peut agir sur le contenu des lois de finances en modifiant la loi organique qui les régit. Il est donc insatisfaisant que le Gouvernement n'ait pas trouvé le moyen, au cours de ces discussions ô combien nourries, nourries, de faire apparaître dans la loi soumise à notre vote le dispositif de remplacement qu'il avait pourtant annoncé.

Il y a, me semble-t-il, une petite méprise : personne, ici, n'imagine que notre rôle territorial, que la fonction d'accompagnement, de soutien, de conseil

la proposition avancée par le Gouvernement, à la suite des engagements du Président de la République et des délibérations de nos deux assemblées, est largement positif. C'est ce qui me conduit à observer, avec un certain sourire, qu'après tant de protestations nous allons voter très massivement pour ce projet de loi

Ainsi, les travaux de l'Assemblée nationale se sont déroulés hier ! Comment pouvons-nous examiner ce projet de loi organique dans de telles conditions, alors même que de nombreux articles restent en discussion- seuls cinq articles ont été adoptés de manière conforme ? Comment exercer notre droit d'amendement, légitime et inaliénable ? Il est vraiment désolant de constater, chez les promoteurs d'un monde nouveau, ce que j'appelle, en pesant mes mots, un mépris envers le Parlement et ses travaux. Ce mépris, d'ailleurs, est relayé par le nouveau président de l'Assemblée nationale qui appelle, lui, tout simplement, à se passer de la séance publique ou bien à réduire l'examen à une seule lecture par chambre. C'est donc un antiparlementarisme basique

Un thème aussi important que celui de la confiance dans l'action publique aurait mérité un examen approfondi, à la hauteur de la défiance immense qui s'exprime dans notre société, comme nous pouvons le constater à chaque élection.

au coeur de l'été. Croyez-vous réellement rétablir la confiance avec des ordonnances, une pratique qui va précisément à contre-courant de cette restauration de la confiance et de l'exigence de transparence

nous semble très positive. D'autres ont pour objet d'encadrer les activités de conseil développées par les parlementaires, lorsque ces activités sont créées postérieurement à l'exercice du mandat. Nous regrettons, à ce sujet, que les amendements visant une interdiction totale des activités rémunérées pour les parlementaires, ainsi que les amendements tendant à imposer une publicité des clients des cabinets auxquels ces parlementaires étaient rattachés aient tous été refusés. Il est pourtant temps d'en finir, aussi, avec ces pratiques

Il nous semble que nos assemblées gagneraient à plus de diversité et fatalement, ce type de questions sur les rémunérations complémentaires se poserait moins. Il est temps de fermer nos institutions aux forces de l'argent et aux lobbys pour retrouver le sens de l'intérêt général et du bien commun. venons-en au principal point de cette nouvelle lecture : la réserve parlementaire. L'Assemblée nationale s'est prononcée pour une suppression sèche à l'horizon de 2024, tandis que le Sénat préconise un maintien sous une autre forme, plus encadrée, avec une transparence renforcée, adossée à un fléchage plus clair vers les collectivités territoriales. Nous pouvons discuter très longuement de la légitimité qu'ont, ou pas, les parlementaires pour affecter des subventions.

Je tiens à préciser que les membres de mon groupe ont utilisé cette réserve utilement, au bénéfice de l'intérêt général. Donc tout peut s'entendre. Mais sur le fond, aucun des membres du groupe communiste républicain et citoyen ne peut accepter que soit remis en cause l'intérêt de ressources mises au service des territoires, à l'heure où les collectivités territoriales, par conséquent les populations, sont durement touchées par les politiques d'austérité de ce gouvernement dit « du renouveau », mais qui marche au même pas que les précédents. Je rappelle C'est le montant, confirmé lors de la Conférence nationale des territoires, de la nouvelle saignée infligée aux collectivités, qui sont pourtant à l'os. Le Gouvernement enfonce le clou, puisqu'un décret a été pris afin de supprimer 216 millions d'euros dans les crédits de paiement de la mission « Relations avec les collectivités territoriales

que subsiste un flou, madame la ministre, quant à la promesse de sanctuarisation de fonds dédiés dans la prochaine loi de finances à l'automne prochain. En ne s'attaquant pas aux racines de la défiance et de la colère populaires, ce projet de loi organique est une occasion manquée pour rétablir la confiance dans l'action publique et dans la vie politique. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons une nouvelle fois. Comme l'écrit un auteur célèbre pour ses citations, « quand la confiance est absente, la méfiance danse ». Avec ce texte, je crains qu'elle ne danse encore longtemps.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le président-rapporteur, mes chers collègues,

Pourtant ce dimanche, dans l'église de ce petit village, sera raccroché un tableau représentant le baptême du Christ. Classé monument historique, ce tableau croupissait dans le fond de la sacristie dans un état de dégradation avancé.

J'ai choisi cet exemple parmi les dizaines de dossiers de ce type que j'ai traités au cours d'une vie parlementaire certainement trop longue à vos yeux. Qu'il y ait eu des abus dans l'utilisation de cette réserve, c'est probable. Est-il pour autant utile de supprimer ces aides profitant essentiellement aux communes modestes ? Depuis plusieurs années, en rendant publiques les aides accordées, le Sénat a régulé cette utilisation. Le président Philippe Bas avait fait adopter en première lecture un processus encore plus clair et plus contraignant. La majorité de l'Assemblée nationale s'enferre dans un dogmatisme aveugle et consternant. Si seulement le Gouvernement en restait à cette suppression s'y ajoute le coup de rabot annoncé dans les dotations qui vient d'être évoqué à hauteur de 300 millions d'euros. Là encore, ce sont les communes rurales aux budgets étriqués qui en pâtiront prioritairement. Comme le rappelaient certains orateurs mercredi dernier, il convient, outre cette question, de relativiser la portée globale de ce projet de loi organique, après celle du projet de loi adopté mercredi. « L'humilité épargne les affres de l'humiliation », écrivait Georges Bernanos. C'est pourquoi nous serions bien avisés de ramener ces textes à ce qu'ils sont pour l'essentiel, quel que soit leur intitulé final : un agrégat de mesures de colmatage destinées à perfectionner des dispositifs existants. D'une manière plus générale, le Gouvernement reprend les vieilles ritournelles antiparlementaristes et s'inscrit dans la continuité des modifications introduites par les lois de transparence adoptées sous le précédent quinquennat, au lieu de la modernité attendue et promise par le candidat Emmanuel Macron. Il n'est pas question de tourner le dos aux réformes institutionnelles qui s'imposent. Personne d'entre nous n'ignore qu'elles sont nécessaires pour redonner de la vitalité à notre régime démocratique. En seize années de présence à la Haute Assemblée, j'ai été témoin de sa capacité réformatrice, quand ses propositions ne sont pas ignorées par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement. Sur des sujets aussi importants, par exemple le phénomène de pantouflage des hauts fonctionnaires, la précipitation induite par le recours à la procédure accélérée n'est pas de nature à instaurer un climat d'examen serein, comme Mme Assassi

Le Gouvernement en est pour partie responsable, en raison de son refus d'approfondir les sujets soulevés par les parlementaires. Je considère pour ma part que la prévention des conflits d'intérêts aurait mérité des mesures plus rigoureuses que le système d'incompatibilité relative avec les activités de conseil ici proposé. De l'ambiguïté découle souvent l'affaiblissement de l'autorité. Malgré ces regrets, je tiens à saluer le travail des membres de la commission mixte paritaire destiné à instaurer un meilleur parallélisme entre les règles s'imposant au législatif et à l'exécutif. Il n'était pas acceptable que les exigences de probité et de moralité imposées aux membres du Gouvernement diffèrent de celles qui échoient aux parlementaires. La grande majorité des membres du groupe du RDSE soutient également les efforts entrepris pour préserver l'aide financière des parlementaires aux petites collectivités. Il serait en effet paradoxal de supprimer un outil budgétaire devenu transparent, qui permet de soutenir l'investissement au niveau local avec une grande réactivité au moment où l'on condamne la lourdeur administrative et où les dérives observées concernent uniquement les dépenses de fonctionnement des collectivités. À ce stade des discussions, je continue de penser que la suppression catégorique de la réserve parlementaire serait une erreur. ces textes porteront-ils leurs fruits à long terme. C'est une question que l'on peut se poser. Pour l'heure, ils semblent avoir surtout donné lieu à la réactivation de crispations et à des prises de position caricaturales. Certains voudraient faire de l'adoption de ce projet de loi organique un moment de bascule entre un « ancien monde » et un « nouveau monde » politique. Mon expérience législative m'a néanmoins permis de constater que les transformations s'inscrivent dans le temps long, et qu'il ne faut pas confondre l'écume des lois et les marées législatives, pour reprendre une image chère à Fernand Braudel. L'antiparlementarisme ambiant agité par certains médias et que le Gouvernement entend relayer ne peut que nous faire craindre un jour ou l'autre le triomphe des extrêmes. En quinze ans, le taux d'abstention au second tour des élections législatives a augmenté de près de vingt points, passant de 39,7 % à 56,4 %. Il est incontestable que la lutte contre ce phénomène doit demeurer une priorité après l'adoption de ce texte, adoption qu'une majorité des membres du groupe du RDSE et moi-même soutiendrons, compte tenu des améliorations introduites par la Haute Assemblée. La parole

le Sénat parvient aujourd'hui au dernier stade d'un débat qui était attendu de longue date par nos concitoyens, celui qui concerne le rétablissement de la confiance dans les structures fondant notre vie démocratique. Ce débat était un engagement de campagne du Président de la République. C'était aussi, et surtout, une nécessité après les innombrables polémiques nées au cours de la campagne électorale. La Haute Assemblée a cherché, depuis près de deux mois, à travailler dans un esprit d'ouverture et de dialogue avec le Gouvernement et la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Notre objectif n'a jamais dévié : déterminer le meilleur équilibre possible entre les intentions initiales du Gouvernement et les réalités de l'action publique. Le groupe Union Centriste du Sénat, que je représente aujourd'hui, se félicite de constater que, après la commission mixte paritaire de mardi dernier, nos convergences ont permis de définir un texte commun concernant la loi ordinaire, désormais en attente de promulgation.

Sur ce sujet, on le sait, il y a pu avoir des dérives par le passé. Néanmoins, l'idée que la réserve soit une bourse à la corruption des grands électeurs est un mythe.

Sur le plan de la méthode, je ne peux que regretter l'attitude qui nous a été décrite de Mme la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de la commission mixte paritaire de mardi. Déclarer que le Gouvernement ne veut pas de la réserve sous quelque forme que ce soit ne tient pas lieu d'argument suffisant. Je déplore, ainsi que mes collègues du groupe de l'Union Centriste, que le débat lors de la commission mixte paritaire n'ait pu être à la hauteur des enjeux, de sorte que j'espère que vous pourrez, madame la garde des sceaux, nous renseigner sur les raisons justifiant cette obstination, malgré les travaux du Sénat, de la majorité des groupes politiques et de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Sur le fond du dossier, je souhaite rétablir une fois pour toutes quelques vérités au bénéfice de nos concitoyens. La réserve parlementaire n'est pas un instrument de népotisme. Aucun parlementaire ne se promène, même le dimanche, dans son territoire d'élection un carnet de chèques à la main. La réserve est en revanche le seul outil d'intervention directe à la disposition du parlementaire. C'est un outil modeste : 146 millions d'euros répartis entre plus de 900 parlementaires.

Combien d'églises ou d'autres monuments essentiels de notre patrimoine local ont été sauvés grâce à la réserve ? Nul ne saurait le dire tant ces crédits jouent un rôle important pour assurer le lien entre le travail du parlementaire et la vie locale réelle., réelle., des efforts notables ont été réalisés depuis plusieurs années pour garantir la transparence de la réserve. Les crédits sont consultables en ligne et il est de plus en plus fréquent que les parlementaires- c'est mon cas -fassent eux-mêmes la publicité de leur engagement dans tel ou tel projet local au moyen de la réserve. La suppression de la réserve pose également un problème démocratique majeur. Comment expliquer que l'on supprime un levier financier d'action à des responsables politiques démocratiquement élus, alors que l'on confie l'opportunité de la ventilation de la le FSIL, à des préfets, des préfets de région, c'est-à-dire des fonctionnaires nommés par l'exécutif et qui n'ont à répondre qu'auprès de lui ? Si c'est cela le rétablissement de la confiance, cela en dit long sur la suspicion que

9, tel qu'il est rédigé, n'est rattachable à aucune disposition constitutionnelle clairement identifiée et justifiant l'intervention du législateur organique., interdire une pratique qui n'est jamais définie ne me semble pas être un exercice de bonne législation. Le Conseil constitutionnel devra nécessairement se prononcer sur ce point du texte et cet aspect du débat devrait nous pousser à nous engager tous autant que nous sommes dans un débat de fond sur les voies et moyens permettant de sauvegarder une forme de réserve parlementaire rénovée, encore plus transparente et au service de l'investissement local et des associations. La solution proposée par le Sénat et revue par la commission des finances de l'Assemblée nationale permettait de répondre au besoin de soutien financier des collectivités et des associations.

Dans ces conditions, et en associant mon collègue Yves Détraigne à mes propos, je crois fermement que notre débat de cet après-midi peut nous permettre de définir un compromis rendant possible de concilier votre intention, madame la garde des sceaux, avec nos impératifs. Nous avons trouvé une solution commune sur les modalités de prise en charge des frais de mandat ; nous avons trouvé une solution pour endiguer la pratique des emplois familiaux ; nous avons commencé à élaborer un statut législatif du collaborateur parlementaire.

Au-delà, madame la garde des sceaux, le débat de ce jour n'a pas vocation à clore, au Sénat, le travail sur la réforme institutionnelle, qui prendra la forme d'une révision constitutionnelle pendant la prochaine session ordinaire du Parlement. nous sommes aujourd'hui seulement en train de poser la première pierre d'un édifice qui a besoin de solides fondations pour durer. Je ne doute pas qu'à l'orée de cet important cycle de travail qui est devant nous, vous saurez, dans ce débat, faire preuve d'écoute, d'ouverture et de dialogue. La parole

Les situations politiques peuvent conduire à ce que les deux chambres constatent des désaccords entre elles. Les positions sont exprimées, les arguments sont échangés et c'est le rôle de la commission mixte paritaire d'en prendre acte.

» ! Alors que nous leur demandions d'échanger avec nous sur nos arguments, nous n'avons obtenu aucune réponse. On comprend qu'ils n'aient pas envie de changer d'avis,

loi organique de Bruno Le Roux, votée à l'Assemblée nationale au mois de février 2017, mériterait toute notre attention et une reprise par le Gouvernement. Elle précise les obligations déclaratives et déontologiques des membres du Conseil constitutionnel qui,

La réserve parlementaire n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elle était au cours des années 2000 et avec la pratique de cette époque. Absolument ! Depuis 2011, l'exigence de transparence et d'équité a été entendue. Ce qui était auparavant un scandale- de l'argent public distribué sans transparence par des parlementaires aux enveloppes très variables -est devenu transparent et normé. Cette victoire de la transparence, nous la devons aux élus qui, depuis 2011, ont travaillé sur ce sujet et aussi aux citoyens qui se sont battus pour cela. La confiance, madame la garde des sceaux, ne se décrète pas ; elle se construit progressivement en faisant les bonnes choses au bon moment et en expliquant ce qui est possible et ce qui ne l'est pas.

d'être rappelé : « Il est mis fin à la pratique dite de la réserve parlementaire » consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées. relative aux lois de finances l'obligation de publication des subventions attribuées sur proposition du Parlement. Quel est le fondement en droit de la réserve aujourd'hui ?

qu'il ne dépose pas d'amendement lors de la discussion budgétaire et le dossier est clos ; si le Parlement ne veut plus de la réserve, qu'il ne vote pas l'amendement du Gouvernement et le dossier est également clos. C'est tout simple et c'est la seule solution en droit. Pourquoi diable vouloir limiter le pouvoir d'amendement du Gouvernement

Que penser d'une loi organique qui limite la liberté constitutionnelle d'amendement du Gouvernement ? Lors du débat à l'Assemblée nationale, madame la garde des sceaux- vous l'avez souligné tout à l'heure -, certains ont expliqué que la pratique de la réserve parlementaire était anticonstitutionnelle.

un amendement et a ainsi amélioré encore la pratique de la réserve. On pourrait aller encore plus loin en menant un débat constructif, plutôt que ce non-débat avec l'Assemblée nationale.

Comment peut-on faire ? Face à ces annulations de crédits et aux enjeux que cela représente pour les départements ministériels concernés, les 146 millions

parce que nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que l'ensemble des actions soutenues par la réserve ne puissent plus disposer d'un soutien financier public. Ce soutien construisait un lien de confiance dans l'action publique, dans ceux qui la conduisent ; il témoignait notre connaissance des réalités de terrain et c'est ce lien que nous cassons.

je voudrais en quelques observations, madame le garde des sceaux, vous dire pourquoi vos explications ne nous ont pas convaincus. Je ferai une observation d'ordre général et deux observations plus spécifiques sur la fameuse réserve parlementaire. D'abord, une observation d'ordre la confiance ne se décrète pas, et, vous le savez bien, il faudra beaucoup plus qu'un texte pour la rétablir.

Franchement ! Nous parviendrons à rétablir la confiance dans la vie politique quand la politique commencera à obtenir des résultats concrets pour la vie des Français en matière de chômage, de pouvoir d'achat,

En réalité, derrière cette intransigeance et derrière nos différences, il y a de vraies divergences : une divergence sur la conception que nous nous faisons du rôle des élus- y compris des parlementaires -et une divergence sur le rôle que nous

comme si cette position exprimait une vision de la politique, ou plutôt de la sortie de la politique, réduite à une forme de rêve technocratique finalement, la fin du clivage serait simplement la réduction de la politique à ce qu'on pourrait appeler une fonction uniquement administrative des choses de la cité. « L'administration des choses plutôt que le gouvernement des hommes

nous permettent d'y voir plus clair sur le rôle que vous voulez attribuer aux élus, qui sont des corps intermédiaires importants et que vous pourriez affaiblir.

Paris n'a d'yeux que pour l'intérieur du périphérique et que, au-delà, la France n'existe pas. Eh bien, ces territoires disposeront de moins de moyens pour assumer la charge des services publics, de l'investissement public qu'ils doivent à leur population.

plus personne ne l'ignore, la commission mixte paritaire, réunie mardi dernier, n'a pas été en mesure de trouver un accord sur ce projet de loi organique. Cette absence d'accord illustre des approches radicalement différentes des deux assemblées qui ont examiné ce texte. Les choses avaient pourtant bien commencé, et l'on ne dira jamais assez combien le patient travail de notre président-rapporteur a permis de faire adopter par l'Assemblée nationale un grand nombre de dispositions ambitieuses introduites par le Sénat dans le projet de loi ordinaire. partis d'un texte lacunaire, qui témoignait d'une volonté insidieuse d'introduire le soupçon- du moins le doute -à l'égard des élus. Le contenu du texte était fort éloigné d'une conception de l'éthique qui s'imposerait à l'ensemble des acteurs de la vie publique. Le Sénat a permis de rééquilibrer le projet de loi ordinaire, afin de concilier la nécessité de la transparence de la vie publique et le respect des droits et libertés fondamentaux. En revanche, s'agissant du projet de loi organique, la commission mixte paritaire n'est pas parvenue au même résultat, en raison essentiellement d'un profond désaccord sur la suppression de la réserve dite « parlementaire Je regrette profondément que ni l'Assemblée nationale ni le Gouvernement n'aient souhaité entendre la voix de nos collectivités territoriales. Tout d'abord, j'aimerais rappeler quelques réalités sur ce dispositif que l'on appelle la « « réserve parlementaire ». Que n'a-t-on dit à son sujet, entre approximations, balivernes et fantasmagories ? Contrairement à ce qui a été affirmé dans les médias et dans le discours du Gouvernement, la dotation d'action parlementaire n'est pas une somme d'argent distribuée arbitrairement par un parlementaire. Il s'agit de crédits inscrits en loi de finances, essentiellement au bénéfice de projets d'investissement locaux, comprenant des pièces de dossier instruites et contrôlées par le ministère de l'intérieur et par les préfectures. Ce n'est donc pas une manne insaisissable et floue que chacun répandrait et dilapiderait selon son humeur et sa prodigalité. Au contraire, ce sont souvent des aides qui peuvent se révéler essentielles pour des projets d'investissement de petites communes qui n'auraient pas eu d'appui financier autrement.

Chacun y trouvera des projets d'accessibilité pour les personnes handicapées, de préservation du patrimoine culturel ou de rénovation de crèches. On dira que c'est une liste baroque ou un inventaire à la Prévert. Il n'y a cependant rien de dégradant ou d'infamant à participer à faire émerger de tels projets, importants pour des territoires ruraux souvent oubliés. Le Sénat s'est toutefois montré prêt à travailler avec le Gouvernement. Nous avions élaboré un dispositif alternatif répondant aux exigences de transparence et préservant, en même temps, les ressources des collectivités locales. Nous avions proposé la création d'un fonds de soutien à l'investissement réservé aux communes et à leurs groupements, renforçant les garanties en matière de transparence, avec des critères d'éligibilité. Nous avions proposé la participation de droit de tous les parlementaires aux commissions attribuant la DETR. Nous avions aussi renforcé les exigences de publicité s'agissant de la réserve dite ministérielle, avec une publication annuelle en. La La chronique parlementaire retiendra que le Sénat s'est montré prêt à renforcer les exigences de transparence dans l'attribution de ces fonds tout en proposant un dispositif alternatif sécurisant les ressources des communes et sanctuarisant une dotation de solidarité.

dont l'État est le premier et principal auteur. Cette situation est particulièrement déresponsabilisante. En trois ans, c'est une ponction de 11 milliards d'euros qui a été réalisée sur les budgets locaux. Pour les cinq prochaines années, c'est une réduction de 13 milliards d'euros qui a été annoncée, laquelle s'ajouteront la suppression de la taxe d'habitation et le gel de 80 % des crédits destinés à l'équipement des territoires ruraux et au soutien à l'investissement local. C'est un camouflet aux 500 000 élus locaux, bénévoles pour la plupart, que vous allez achever de décourager, alors même qu'ils mesurent chaque jour la nocivité de la loi NOTRe et ses funestes conséquences. Madame la ministre, comment voulez-vous que le Sénat, représentant des collectivités locales, accepte de supprimer ce levier de développement local en direction de multiples petits projets ? Le Gouvernement et sa majorité sont restés engoncés dans leurs certitudes et ont soigneusement évité de rechercher une alternative à cette suppression pure et simple. Et que dire de l'attitude des députés membres de la commission mixte paritaire qui ont mécaniquement

Je dis « totem », car, pour mettre fin à cette pratique, il suffisait au Gouvernement de ne pas déposer d'amendement abondant la ligne budgétaire au moment de la prochaine loi de finances. Mais vous avez recherché à tout prix, sur fond déclamatoire pour mieux le brandir, un symbole plutôt qu'une analyse proportionnée et raisonnable, manifestant par là une forme d'infantilisme dans cette préférence donnée à l'affichage des bonnes intentions, au détriment de l'amélioration d'instruments et d'outils de développement local. Je dis « infantilisme », car je ne peux m'empêcher de penser à Milan Kundera, qui disait que la maturité, politique en l'espèce, se mesure à la capacité à résister au symbole.

représente les collectivités locales ne puisse suivre l'Assemblée nationale sur un chemin aussi hasardeux qu'incertain. Elle revotera donc le texte proposé par notre président-rapporteur, qui aurait dû vous inspirer bien plus fortement. La discussion

conserver la faculté de faire appel à des parlementaires pour la conduite de missions diverses afin d'enrichir sa vision sur de nombreux sujets, comme ce fut le cas ces dernières années pour la simplification ou la propriété intellectuelle. Ces travaux ont fréquemment lieu en amont du processus législatif et peuvent associer des compétences et des profils variés, issus de l'administration centrale, des inspections générales, du Conseil d'État, et également d'institutions comme la Cour des comptes qui sont indépendantes du pouvoir exécutif. Ils nourrissent aussi la réflexion du Parlement

à laquelle vous nous avez habitués vous retiriez votre amendement, ce qui signifierait au moins que, sur le plan des principes, vous êtes d'accord avec nous et considérez qu'il vaut mieux mettre un terme à une pratique malsaine. La parole Madame la ministre,

mais je vous assure que la disposition votée par la commission a été correctement rédigée. La référence à l'article que vous avez cité est exacte : elle concerne les sénateurs et entrera en vigueur prochainement.

ou on modifiait des lois ; voilà maintenant qu'on abroge des pratiques, une coutume ! Étrange innovation, étrange perversion juridique ... Madame la garde des sceaux, votre majorité serait-elle saisie par un nouveau virus, celui de l'inconstitutionnalité ? Sur le fond, si l'on supprime purement et simplement la réserve parlementaire comme le prévoit l'article 9 tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, encore faudrait-il trouver un mécanisme de substitution. Le président de notre commission des lois, M. Philippe Bas, a trouvé une excellente formule qui associe les élus au maintien de subventions aux petites communes et aux besoins d'investissement des Français de l'étranger. La majorité à l'Assemblée nationale continue à s'opposer à ce dispositif performant. Cela suscite de légitimes inquiétudes chez tous nos collègues représentant les Français de l'étranger, parlementaires et conseillers consulaires, car nous serons doublement impactés, n'ayant pas de collectivité territoriale pour nous venir en aide. À voir ce qui se passe pour les collectivités territoriales, l'État risque de ne pas compenser cette suppression en période de vaches maigres, où le rabot de Bercy- ce n'est pas un verrou, mais un rabot permanent -fonctionne énergiquement dans tous les ministères, à commencer par celui de l'Europe et des affaires étrangères. D'abondantes suppressions de crédits y sont annoncées. Une grande partie des restrictions devraient concerner l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et donc nos établissements scolaires. Madame la ministre, vous avez pris des engagements à l'Assemblée nationale. Permettez-moi de reprendre vos propos : « Je le dis très clairement et je m'engage sur ce point-là : il ne faut pas que les bénéficiaires des fonds qui aujourd'hui transitent par la réserve soient lésés. « Il n'est pas question de faire des économies sur le dos des collectivités, des Français de l'étranger et des associations, dont nous connaissons évidemment tous ici le rôle essentiel. « Pour tous ces bénéficiaires, le Gouvernement est sensibilisé et trouvera les solutions adaptées d'ici au prochain projet projet de loi de finances. » Madame la ministre, s'il faut en croire vos déclarations, les Français de l'étranger et les communes rurales vont avoir un avenir ensoleillé. En êtes-vous sûre ? Quand vous parlez des dispositifs existants qui permettront de récupérer une partie des sommes confisquées par la suppression de la réserve, vous évoquez des aides aux collectivités territoriales et aux associations oeuvrant en France ... Mais, les Français de l'étranger, où sont-ils dans votre raisonnement ? Comptez sur toute ma vigilance pour qu'ils ne soient pas les sempiternels oubliés. Je vous avoue que j'attends, avec mes collègues représentant les Français de l'étranger comme avec mes collègues sénateurs représentant les communes rurales, oui, j'attends avec une impatience non dissimulée la parution du projet de loi de finances, qui nous amènera certainement à revenir vers vous.

qu'ils soient en investissement pour les collectivités locales ou en fonctionnement pour les associations ? Nous ne manquerons pas de renvoyer la

vous vous méprenez complètement sur les conséquences en termes d'emploi. On pourrait imaginer que ce sont les parlementaires qui distribuent des liasses. Mais ce n'est pas

de nombreuses alliances françaises allaient mettre la clef sous la porte, et pour cause : la plupart d'entre elles vivent des subventions qu'elles peuvent recevoir au titre de la réserve parlementaire.

les 1, 2 million d'euros dont j'ai disposé au titre de la réserve parlementaire depuis que je suis élu, plus de 600 000 euros ont été destinés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,

Je sais la satisfaction des bénéficiaires. Je sais ce qu'ils ressentent quand on leur donne de quoi terminer un projet, par exemple

et plus claire, ... Non ! ... raison pour laquelle je m'évertue à en faire devant vous la démonstration. Ces deux logiques sont tellement différentes

d'apporter des restrictions au droit d'amendement du Gouvernement. Il me semble qu'il y a là une erreur d'analyse. L'article 44 de notre Constitution le précise clairement : c'est une loi organique qui fixe le cadre du droit d'amendement,

dans une grande ville, certes, mais nous avions une politique de subventions pour les petites associations, et je puis vous assurer qu'il nous arrivait de donner de petites sommes pour des festivals modestes. Cela aussi fait partie des choix politiques que nous avons à faire.

Nous sommes animés, vous, moi et l'ensemble de cette assemblée, par une égale aversion envers toute démagogie. Mais qu'est-ce que la démagogie ?

l'accès des communes rurales et celui des associations de Français de l'étranger à des financements, ils ne s'expriment pas de manière démagogique. Ils s'expriment de manière pragmatique et réaliste. Très bien ! Ils n'ont pas échafaudé une théorie sur la mission des parlementaires,

permis de remédier à l'impossibilité constatée d'un accès à la ressource publique pour ces petits projets qui sont hors du champ de vision de l'État.

paritaire étaient bien à la recherche d'un consensus sur cette question délicate. Nous ne sommes donc pas dans le cas de figure qui a été tranché par le Conseil constitutionnel dans une décision de 2015, mais dans une tout autre situation : celle où un accord était souhaité, et où la recherche de cet accord, qui passait par un vote, a été refusée par le président de la commission mixte paritaire. Le Conseil constitutionnel aura à apprécier si la Constitution a été respectée sur ce point de procédure, qui nous paraît tout à fait essentiel.

à la constitutionnalité de cette disposition. Supposons que l'on puisse l'interpréter comme une restriction au droit d'amendement du Gouvernement. Vous connaissez mieux que moi la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment la décision du 25 juin 2009. L'article 44 de la Constitution, que vous invoquez pour dire que la loi organique pourrait restreindre le droit d'amendement du Gouvernement ou du Parlement, ne me paraît pas pertinent. cet article se borne à indiquer, en renvoyant d'ailleurs tant au règlement de chacune des assemblées qu'à la loi organique, que c'est à ces deux instruments de préciser les conditions d'exercice du droit d'amendement. Quant aux restrictions au droit d'amendement, il va de soi

appliquer soit l'article 40, sur les irrecevabilités financières, soit l'article 41, sur les irrecevabilités résultant du partage entre la loi et le règlement, soit l'article 45, qui a fait l'objet d'une abondante jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce que l'on appelle les « cavaliers législatifs » et la fameuse règle « de l'entonnoir », métaphores qui nous sont devenues familières ... Nous sommes alors en présence d'un véritable fondement constitutionnel des restrictions à l'exercice du droit d'amendement. Pas avec l'article 44 de la Constitution ! La loi organique ne peut en aucun cas restreindre

le Conseil constitutionnel a fait le ménage parmi les neutrons législatifs. Lorsqu'il estime que telle disposition d'une loi organique ou d'une loi ordinaire n'a pas de fondement dans la norme supérieure et n'énonce aucune

dans le projet de loi organique qu'il nous présentait. Il n'a pas été possible d'obtenir satisfaction sur ce point. Vous aurez donc l'éphémère satisfaction d'obtenir de l'Assemblée nationale ce que vous voulez en obtenir, madame la ministre. Le Conseil constitutionnel ne l'entendra certainement pas de cette oreille madame la ministre.

Le scrutin est ouvert.

dans le texte de la commission, l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé

Le scrutin est ouvert.

M. le président du Sénat prendra acte de la clôture de cette session lorsque nous aurons reçu le décret de M. le Président de la République Sauf élément nouveau, le Sénat se réunira le lundi 2 octobre 2017, à quinze heures, avec l'ordre du jour suivant : Installation du bureau d'âge. Ouverture de la session ordinaire 2017-2018. Allocution du président d'âge. Scrutin secret à la tribune pour l'élection du président du Sénat. Fixation du calendrier de la suite du renouvellement des instances du Sénat. Je souhaite d'excellentes vacances à tous ! Personne ne demande la parole ? ... La séance est levée.